La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

Cet amendement est de bon aloi, car il a été proposé par Jacques Toubon, Défenseur des droits,

Le second est de préciser que, en cas de doute sur l'authenticité des documents, le doute bénéficie au demandeur de la réunification familiale. Ce dernier point est évidemment très discutable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. D'abord, la définition des liens de filiation est très complexe. Il convient de laisser aux services le soin de l'apprécier. En outre, il faut rappeler que les consulats peuvent également consulter le registre d'état civil du pays d'origine et demander des informations à l'OFPRA. C'est évidemment prévu dans le CESEDA.

si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dans ces conditions, et compte tenu de la fraude rencontrée massivement- je dis bien : massivement -dans certains pays d'origine, le Gouvernement est défavorable au fait d'ériger en principe une présomption, même simple, de sincérité donnée à des documents douteux. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable

Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen porte exclusivement sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Il s'agit d'assurer que l'examen médical ait un lien direct avec la demande de protection. Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite « directive Procédures dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires, sous réserve du consentement du demandeur, pour que celui-ci soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.

Lorsque l'OFPRA demande au demandeur d'asile de réaliser un examen médical, c'est parce qu'il lui est nécessaire pour mener à bien sa mission de protection. Par exemple, lorsque cet examen concerne une jeune fille protégée contre un risque d'excision- elle n'est donc pas excisée -, il est contre-productif de demander qu'il ne porte que sur les atteintes subies par la personne. Cela priverait la protection de sa portée. Un examen médical peut en effet être indispensable afin de mieux évaluer, de mieux identifier les craintes de persécutions et d'atteintes graves de ces personnes à la lumière des éléments de la demande d'asile. Il ne s'agit en aucun cas de demander un examen à des fins autres que celles de protection ou d'exercer un quelconque contrôle. À cet égard, la précision que vous souhaitez apporter ne nous paraît absolument pas utile. Le Gouvernement demande donc le

Procédures du 26 juin 2013, que j'ai citée précédemment, les États membres prennent « les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé ». À défaut d'examen médical, l'alinéa 2 du même article

-de prévenir le demandeur qu'il peut réaliser un tel examen, d'autant plus que le certificat médical, en cas de séquelles physiques, mais aussi psychologiques, peut se révéler être une pièce essentielle du dossier,

Préciser qu'il peut être informé d'une telle possibilité, outre le fait que cela ne relève pas du domaine de la loi, ne paraît donc pas nécessaire. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Autrement, l'avis sera défavorable. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

importante. Il est toujours envisageable, même si, bien évidemment, l'OFPRA fait parfaitement son travail, qu'à un moment ou à un autre un examen médical n'ait pas été mené l'un des problèmes soulevés par le demandeur, ne serait-ce que parce que celui-ci, nous y reviendrons tout à l'heure, ne s'est pas exprimé dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Dans ces conditions, il paraît opportun que le demandeur puisse à son tour, conformément à la directive, demander qu'un examen complémentaire soit réalisé, même si c'est effectivement à lui de le financer.

Le scrutin est ouvert.

avant la fin de la procédure ne puissent pas bénéficier de la réunification familiale. Une telle modification va à l'encontre du droit d'asile et du droit à vivre dans une famille réunifiée. Par conséquent, nous ne pouvons faire autrement que de voter contre l'article

Cela devrait aller de soi, mais ni la convention de Genève ni la directive Qualification ne les mentionnent expressément. La convention de Genève évoque, dans son article 1, les persécutions « du fait de [la] race, de [la] religion, de [la] nationalité, de [l'] appartenance à un certain groupe social ou [des] opinions politiques ». La directive Qualification, quant à elle, mentionne, dans son article 10, au titre des motifs de persécution, la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques ». Par conséquent, les aspects liés au sexe, pourtant

les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. L'amendement que nous défendons a pour objet de préciser la liste des traits pouvant faire l'objet de persécutions, en y ajoutant la question de l'identité de genre. En effet, nous ne pouvons ignorer la question de la transidentité et les difficultés qui sont celles des personnes transgenres dans certains États menant une politique de répression Nous ne pouvons pas non plus ignorer la difficulté qui est la leur au sein de nos centres d'accueil et de rétention administrative, où elles n'ont parfois pas accès à leurs médicaments lorsqu'elles sont en cours de transition,

dans la directive 2011/95/UE traitant des conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

La notion d'appartenance à un groupe social, tel que la prévoit la convention de Genève en son article 1, constitue l'un des motifs de persécution susceptibles d'être pris en compte pour l'octroi du statut de réfugié. L'article 10 de la directive Qualification précise notamment, s'agissant du groupe social, qu'il réunit des membres partageant « une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée », formant un groupe ayant une « identité propre [ ...] parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante ».

n° 119 rectifié. Celui-ci tend à intégrer, au sein des motifs de persécution, les aspects liés à la transidentité, en ajoutant la notion d'identité de genre à celle de genre, qui est déjà prévue dans les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA. conséquent d'ores et déjà satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit que « les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ».

où il existe des motifs sérieux de sécurité, les possibilités pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de refuser ou retirer le statut de réfugié. Il vise également à renforcer l'obligation faite à l'autorité judiciaire de communiquer à l'OFPRA toute information susceptible de justifier une telle décision et, en parallèle, à permettre de procéder à des enquêtes administratives pouvant conduire au refus ou au retrait d'un titre de séjour ou d'une protection internationale. Ici encore, il est proposé de revenir sur les dispositions l'article L. 711-6 du CESEDA, dont la création remonte à moins de trois ans, et ce naturellement pour les durcir, notre commission des lois ayant même souhaité étendre le champ des comportements susceptibles de fonder un refus ou un retrait du statut de réfugié. Des milliers de personnes meurent de vouloir rejoindre le continent européen. Le Parlement et l'exécutif préfèrent au fait d'assurer un accueil digne envoyer un message plutôt plutôt sécuritaire. Rien de surprenant peut-être, mes chers collègues, mais il y a quelque chose de terrifiant à voir des thèses et des idées insidieuses, habituellement réservées à l'extrême droite, aujourd'hui utilisées par par presque tous les bords politiques. Faire penser aux citoyens, qui pourraient être à raison choqués de voir comment la supposée patrie des droits humains traite les exilés, que, parmi ces derniers, se cachent sans doute des terroristes voilà ce contre quoi nous nous battons. Les procédures existent pour refuser ou retirer le statut de réfugié. C'est tout à fait légitime. Mais les durcir nous paraît pour le moins inutile

et de le contraindre à retirer ou à rejeter systématiquement la protection à une personne condamnée à l'étranger pour terrorisme ou pour une infraction punie de plus de dix ans d'emprisonnement. Si l'objectif recherché nous paraît légitime, la rédaction proposée par le rapporteur ne nous semble pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'article L. 711-6 du CESEDA offre déjà un fondement à l'OFPRA pour rejeter une demande d'asile ou y mettre fin, quand la présence de la personne sur le sol français représente une menace grave pour la sûreté de l'État ou lorsque celle-ci a déjà été condamnée pour un crime ou délit puni de plus de dix ans d'emprisonnement. L'automaticité ainsi introduite n'est pas souhaitable. Ensuite, la nouvelle rédaction proposée tend à transformer le rôle assigné à l'OFPRA, en l'insérant dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Cela pourrait nuire à son indépendance, consacrée par l'article 7 de la loi sur l'asile de 2015, qui dispose en effet que l'Office « exerce en toute impartialité » ses missions « et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction Il serait préférable de renforcer à cette fin le contrôle effectué en préfecture, où le personnel est plus familier des questions de sécurité et d'ordre public, et ce dès la phase initiale de la demande d'asile. la rédaction proposée est insatisfaisante, dès lors qu'elle renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation d'une liste des États démocratiques garantissant l'indépendance des juridictions répressives soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Une telle qualification est éminemment politique, comme l'a montré la récente condamnation de Mélina Boughedir en Irak. Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 711-6 du CESEDA, afin d'élargir le fondement d'un rejet ou d'un retrait d'une protection à une personne représentant une menace, en conservant toutefois une marge d'appréciation pour l'OFPRA. également eu le souci de conférer à cet office des moyens utiles dans son appréciation et souhaité maintenir la possibilité, pour les officiers de protection, de consulter certains fichiers administratifs.

dans un État de l'Union européenne ou dans un État tiers pour le refus ou le retrait du statut de réfugié, ce qui pose tout de même une difficulté assez sérieuse. L'amendement tend également à supprimer plusieurs autres apports de la commission, notamment sur la compétence liée de l'OFPRA pour le retrait de la protection subsidiaire. Lorsque l'OFPRA, après

Le scrutin est ouvert.

admiratifs ! Nous constatons toutefois une forme de blocage dans la fluidité de nos débats. En conséquence, monsieur le président,

Le présent amendement vise à modifier l'article L. 711-1 du CESEDA qui dispose que la qualité de réfugié est accordée à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté,

». Nous souhaitons préciser que les militants en faveur de l'égalité devraient également se voir attribuer le statut de réfugié, lorsque leur lutte politique engendre une persécution dans leurs pays d'origine. Valeur cardinale, fondatrice et inaliénable de notre République, l'égalité ne saurait être ignorée dans l'attribution du statut de réfugié. Il y va du respect de nos valeurs comme du droit international et européen. En effet, tant la convention de Genève que la directive 2011/95 de l'Union européenne traitant des conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour bénéficier de la protection internationale ou subsidiaire considèrent que l'opinion politique et donc, de ce fait, la lutte pour les droits civiques et pour l'égalité légitiment une demande de droit d'asile et l'octroi du statut de réfugié, afin de mettre les militants politiques à l'abri des persécutions qu'ils pourraient subir dans leurs pays d'origine. Quel

qui dispose que la qualité de réfugié est accordée à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, en ajoutant qu'elle l'est également si son action est en faveur de l'égalité. Il s'agit ici de modifier l'asile constitutionnel prévu à l'article 53-1 de la Constitution

: « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État

Il s'agit de distinguer la qualification des faits, pour laquelle l'OFPRA a toute latitude dans le cadre de l'instruction des dossiers- sous le contrôle du juge -et la conséquence de cette qualification, qui doit lier l'autorité administrative. L'OFPRA doit ainsi apprécier, premièrement, constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État- c'est donc bien l'OFPRA qui qualifie les faits -, ou, deuxièmement, si le demandeur a été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, si sa présence constitue une menace pour la société française. Les deux conditions sont cumulatives, l'étranger devant nécessairement avoir été condamné définitivement

Le scrutin est ouvert.

à M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement vise à permettre de refuser le statut de réfugié à un demandeur ayant fait l'objet d'une condamnation pour terrorisme en France, dans tout autre État membre de l'Union européenne, partie de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'actuelle rédaction de l'article 4 du projet de loi protège notre pays contre les demandeurs d'asile condamnés pour terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne, mais ne dit rien des autres pays européens. L'Islande, la Norvège, le Liechtenstein ou la Confédération suisse ne sont pas mentionnés dans cet article, alors qu'ils ont noué des partenariats étroits avec l'Union européenne, y compris sur les questions d'asile et d'immigration. Le cas futur du Royaume-Uni est tout aussi important, car, en quittant l'Union européenne,

la rédaction de cet article en interdisant le statut de réfugié aux demandeurs ayant fait l'objet d'une condamnation en France, dans un État membre de l'Union européenne, dans un État membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

à celles prononcées dans un État de l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération helvétique. Il est satisfait par l'alinéa 7 de l'article 4, qui prévoit que sont prises en compte les condamnations prononcées en dernier ressort dans des États tiers, démocratiques et garantissant l'indépendance des juridictions répressives, dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.

le quantum des peines prises en compte dans le refus ou le retrait du statut de réfugié dans la seconde hypothèse de l'article L. 711-6 du CESEDA, lorsqu'il existe des motifs sérieux de sécurité publique. Or cet article constitue la transposition en droit interne de l'article 14 de la directive Qualification, lequel impose de ne prendre en considération que des infractions d'une particulière gravité par leur nature et donc nécessairement punies d'une peine d'un quantum élevé. Abaisser le quantum de la peine risquerait de conduire à méconnaître le sens et la portée de la directive et pourrait nous exposer, en cas de décisions de retrait ou de refus du statut sur ces motifs, à des annulations

Même avis. Ces termes sont effectivement la transposition de l'article 14.4 de la directive européenne dite « Qualification ». Il est souhaitable de faire coïncider au mieux le texte européen et le texte national et de ne pas « abaisser » la

». Je trouve dommageable que, à cause d'un vocabulaire défectueux d'une directive qui ne nous lie en aucune manière en droit, nous écrivions une loi française sur un sujet de cette importance dans un langage qui n'a aucune pertinence.

la communauté que nous formons, des valeurs ? Toutes ces notions, subjectives, n'ont pas place dans un texte de loi. C'est pourquoi nous voterons l'amendement de Mme de la Gontrie. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Roger Karoutchi, pour explication de vote. J'admire, une fois de plus- ça fait beaucoup aujourd'hui -, la capacité d'oubli de certains qui nous font la leçon. Ils semblent ne pas se rappeler le nombre de fois où le groupe socialiste, bien maigrement présent,

Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

amendement tend à préciser que l'appréciation des infractions prises en compte par les dispositions de l'article L. 711-6 du CESEDA pour retirer ou refuser le statut de réfugié en cas de motifs sérieux de sécurité s'effectue au regard du droit national. Sachez que

à l'alinéa 7 de l'article 4. En outre, l'examen auquel se livrera l'OFPRA avant la décision de rejet ou de retrait permettra de vérifier que ces conditions

Cet amendement tend à étendre le refus d'asile aux demandeurs inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, publié en février dernier, compte environ 20 000 personnes selon Matignon,

ce fichier recense exclusivement des individus radicalisés. Mis à jour régulièrement, il permet d'orienter les perquisitions, notamment pendant les périodes d'état d'urgence. Ainsi, les personnes susceptibles de passer à l'acte sont surveillées par la Direction générale de la sécurité intérieure. Les suspects jugés « moins dangereux » sont pour leur part suivis par le Service central du renseignement territorial, tandis que la police judiciaire, les gendarmes et le service de renseignement parisien s'occupent de tous les autres. Il est donc essentiel que ce fichier puisse servir dans l'évaluation d'un dossier de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.

qui permettent de procéder à des enquêtes administratives pour la mise en oeuvre du refus ou du retrait du statut de réfugié pour des motifs sérieux de sécurité publique. Il s'agira d'ailleurs principalement pour l'OFPRA de demander aux services compétents d'effectuer ce qu'on appelle un criblage des individus concernés concernés la consultation des fichiers de police, de justice et de renseignement. L'inscription d'un individu au sein de l'un de ces fichiers- le FSPRT ou le fichier S -sera donc bien prise en compte pour déterminer s'il constitue une menace pour la sécurité publique, la sûreté de l'État ou la société et si

et visant le recueil de renseignements sur des personnes dont certaines peuvent représenter une menace pour l'ordre public, d'autres non. Il ne peut donc fonder une décision de refus automatique, qui, en méconnaissant le principe de proportionnalité, serait contraire à la Constitution et au droit international.

l'amendement proposent que ce refus ne puisse être opposé que si la protection dont bénéficie l'intéressé dans son pays d'origine est effective et non temporaire. qui transpose les termes de l'article 8 de la directive Qualification, dispose que la personne doit être en mesure de s'établir dans ledit pays, ce qui suppose bien que la protection soit effective et non pas temporaire. L'avis est donc défavorable.

pour harmoniser davantage les règles européennes en matière d'asile, la précision que l'amendement tend à apporter serait contraire à l'objectif poursuivi. Elle introduirait au mieux des confusions, au pire des contradictions avec les directives européennes.

Au même titre que les avocats du droit d'asile de l'association ELENA, nous jugeons le présent article incomplet. Aujourd'hui, le refus ou le retrait du statut de réfugié en raison d'une condamnation intervenue dans un État membre de l'Union européenne existe déjà, et ce de manière plus ou moins informelle. Faute d'un encadrement juridique suffisant, les requérants du droit d'asile se voient parfois refuser leur dossier en raison d'une condamnation intervenue dans un pays européen, alors même qu'ils n'ont jamais eu connaissance d'une telle condamnation.

Il s'agit simplement de respecter les droits de la défense, parmi lesquels figure le principe du contradictoire. Pour garantir ce droit, il incombera aux autorités chargées de l'examen des demandes d'asile de faire procéder à la traduction du document relatant la condamnation par un expert assermenté. Dans un État de droit, il apparaît fondamental que le demandeur et/ou son conseil soient avisés de l'existence de cette décision de condamnation et invités à formuler des observations la concernant. Quel est l'avis de la commission

précisément que, lorsque l'OFPRA envisage de mettre fin à une protection, la personne concernée est en mesure de se défendre en lui présentant les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu de lui retirer la protection de lui retirer la protection internationale grâce à une procédure contradictoire. Ainsi, lorsque l'OFPRA informe par écrit la personne concernée des motifs de l'engagement de cette procédure, celle-ci peut présenter par écrit ses observations, et il peut être procédé à un entretien

Éliane Assassi, sur l'article. L'article 5, l'un des plus emblématiques de ce projet de loi, est de ceux qui cristallisent les critiques de l'ensemble des associations et acteurs du droit d'asile. Pour l'essentiel, il réduit le délai de dépôt d'une demande d'asile de 120 à 90 jours à compter de l'entrée sur le territoire afin que celle-ci soit examinée en procédure normale. Ce qui signifie que les demandes déposées après 90 jours seront toutes examinées en procédure accélérée.

l'OFPRA doit, dans ce cadre, statuer en quinze jours, délai qui ne permet pas d'approfondir l'instruction de la demande d'asile. Ce choix va directement à l'encontre des mises en garde de loi par le Défenseur des droits. Celui-ci souligne que, dans un contexte de saturation du dispositif national d'accueil, « rien ne garantit qu'il ne sera pas procédé à des placements injustifiés en procédure accélérée lorsque la personne en quête d'une protection internationale n'aura pas, du fait de la saturation du dispositif, pu déposer sa demande dans le délai imparti, sans toutefois pouvoir justifier de ses tentatives infructueuses ». La possibilité d'accélérer l'examen de la demande est justifiée,

que la directive ne fixe aucun délai maximal au-delà duquel il y aurait lieu de supposer que la demande présente un caractère tardif. Ainsi, le droit interne va sur ce point déjà plus loin que ce qu'exige le droit européen, en prévoyant une présomption de tardiveté pour les demandes déposées au-delà de 120 jours. De plus, cet article réduit ce même délai à 60 jours pour la Guyane, soit un mois de moins que pour la métropole. Nous y reviendrons dans la suite de la discussion, mais le développement du droit d'exception dans le CESEDA est injustifié et fait des territoires ultramarins des territoires de seconde zone. En parallèle, dans le même objectif, cet article dispose que les convocations convocations à l'OFPRA et les décisions de l'Office pourront désormais se faire « par tout moyen », y compris électronique, inévitablement au détriment des demandeurs d'asile, lesquels sont particulièrement vulnérables. Nous reviendrons sur ce point également dans le débat.

le nombre de ces placements. D'un point de vue pratique, en procédure normale, l'OFPRA dispose de six mois pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA de cinq mois après enregistrement du recours. En procédure accélérée, de quinze jours pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA de cinq semaines après enregistrement du recours. De plus, dans ce cas, l'affaire est jugée par un juge unique, non par une formation collégiale. Cette procédure est donc particulièrement désavantageuse pour les demandeurs d'asile. L. 723-6 prévoirait que l'OFPRA puisse convoquer le demandeur d'asile à l'entretien « par tout moyen ». En outre, toutes les décisions de l'Office pourraient être notifiées « par tout moyen garantissant la confidentialité

Un tel élargissement des voies de notification des décisions de l'OFPRA ne va pas, bien sûr, sans poser des difficultés au regard de la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreux demandeurs d'asile, certains sans accès direct à internet, d'autres sans téléphone, entre l'article L. 723-6 permettrait à l'OFPRA d'imposer aux demandeurs d'asile la langue dans laquelle ils seront entendus. En effet, il serait prévu que le migrant peut être entendu dont il a une connaissance suffisante ». Or, selon les associations accompagnant les migrants, il n'est pas rare qu'il soit imposé au demandeur une langue qu'il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en préfecture, alors qu'il cherchait uniquement à manifester sa bonne disposition à l'intégration. Il est très malaisé pour un demandeur dans cette situation de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans son pays d'origine et, plus simplement, de défendre ses droits. C'est pourquoi il est nécessaire, conformément à l'avis du Défenseur des droits, d'abandonner ces dispositions, de même que les alinéas 6 et 7 de l'article 7, par ailleurs contraires à l'esprit de la directive Procédures, puisque les modifications envisagées risquent de compromettre l'accès effectif du demandeur d'asile à la procédure. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l'article. Le placement en procédure accélérée prive tout bonnement le justiciable de la collégialité devant la CNDA et raccourcit le délai de préparation du dossier, au détriment de la qualité de l'instruction. Vous l'aurez compris, nous pouvons ainsi craindre des traitements de dossier à la hâte et, de ce fait, des décisions éthiquement contestables. Par cet article, ce sont les requérants qu'on pénalise dans la formation de leur requête, mais également l'instruction par les agents de la CNDA qu'on dessert, en imposant à ceux-ci une logique de rendement.

individuel « par tout moyen » est injuste. Les rédacteurs du projet de loi méconnaissent-ils la réalité au point de croire que tous les exilés disposent d'un téléphone portable, d'une adresse pour recevoir un courrier postal ou d'internet pour se voir communiquer un Je ne le pense pas. Je crois, hélas, que l'exécutif fait le pari cynique que le nombre de requérants déboutés sera ainsi multiplié, ceux-ci n'ayant pu défendre leur cause, faute de s'être rendus à leur entretien individuel à l'OFPRA. Mes chers collègues, ces exilés qui ont fui la guerre, la misère, les dégradations climatiques ou l'instabilité politique méritent un traitement plus digne de leur demande d'attribution de titre de séjour qu'une procédure déshumanisée et mathématique. La parole est

Je considère en effet qu'il présente un risque d'affaiblissement des droits pour une majorité des demandeurs d'asile. Ainsi, l'abaissement du délai de dépôt d'une demande d'asile

Plus de la moitié des demandeurs d'asile risquent donc de voir leur dossier examiné sous un régime dérogatoire au droit commun, qui présente un risque de prise en compte insuffisante des différentes circonstances éclairant leur situation.

L'article 5 a pour objet la réduction des délais d'instruction des dossiers, actuellement de l'ordre de treize mois. Cet objectif pourrait être partagé, si les services concernés bénéficiaient pour cela de moyens adaptés. est notamment proposé de réduire de 120 à 90 jours le délai à compter de l'entrée sur le territoire au-delà duquel le dépôt d'une demande d'asile peut entraîner l'examen de celle-ci selon la procédure accélérée. Or les moyens choisis pour atteindre ce but consistent exclusivement en une réduction des garanties procédurales, au détriment des demandeurs d'asile : augmentation du nombre de procédures accélérées, réduction des délais de recours devant la CNDA, fin du caractère suspensif de certains de ces recours, choix de la langue de la procédure, convocations envoyées par tout moyen et systématisation de la visioconférence pour les audiences. Les demandeurs d'asile et les professionnels du droit d'asile ont déjà toutes les peines du monde à respecter le délai de 120 jours. Pensez-vous réellement que le délai de 90 jours soit tenable ? La procédure accélérée raccourcit le délai de préparation du dossier, au détriment de la qualité de l'instruction ; elle prive en outre le justiciable de la collégialité devant la CNDA. Toutes ces dispositions méconnaissent manifestement les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par la convention européenne des droits de l'homme.

le demandeur d'asile doit déposer sa demande. La main sur le coeur, on nous affirme que c'est pour réduire les délais d'instruction. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'objectif visé : s'agit-il de protéger au plus vite les demandeurs ou de leur rendre la vie plus difficile et de les décourager, eux et ceux qui seraient tentés, ultérieurement, de choisir la France ? Le Gouvernement n'a pas avancé d'arguments convaincants pour justifier ce recul en matière de délai. En tout cas pas en faisant référence à la directive, qui ne fixe pas de délai limite pour qualifier les demandes Pourquoi revenir sur les 120 jours ? Pourquoi suspecter le demandeur de tarder ? Pour s'installer, pour frauder ? C'est méconnaître la situation des demandeurs. Nombre d'entre nous, à l'occasion de ce projet de loi ou plus souvent, vont à leur rencontre et à celle des associations. Quand on fuit un conflit, qu'on y échappe dans la clandestinité et qu'on est maltraité, voire torturé, par les passeurs ou les autorités des pays de transit, quand on traverse la Méditerranée dans des conditions précaires, qu'on risque de chavirer, qu'on voit ses compagnons de voyage se noyer et qu'on franchit les Alpes en hiver pour échapper aux contrôles, on peut, au moment de penser à sa demande d'asile, avoir besoin d'un temps de répit. Cette semaine, on m'a présenté le cas d'une jeune femme mauritanienne ayant fui son pays du fait d'une menace d'excision. Elle a rejoint en Seine-Maritime sa soeur, qui, elle, n'avait malheureusement pas pu y échapper. Son parcours fut dangereux. Alors qu'elle aurait pu bénéficier d'une protection, elle est restée terrée plusieurs mois chez sa soeur, dépassant les délais, incapable d'affronter les démarches. Des histoires comme celle-là, il y en a des centaines. La plupart des demandeurs ont besoin de temps pour se reconstruire. À cela s'ajoutent la méconnaissance des procédures, la difficulté de comprendre et de se faire comprendre dans une langue maîtrisée, l'isolement, la précarité- 60 % des demandeurs ne sont pas hébergés -et l'absence de conseils, voire de mauvais conseils.

donc rendre précaires leurs conditions d'accès à l'asile.

au demandeur par tout moyen, il s'agit, il est vrai, d'un dispositif nouveau. L'OFPRA a assuré souhaiter mettre en place un dispositif pleinement compatible avec la garantie des droits des usagers.

? Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement, puisque l'article 5 comporte un ensemble de mesures destinées à favoriser la réduction du délai de traitement des demandes, telles que la simplification des modalités de convocation et de notification des décisions

Le choix fait par le Gouvernement semble clair : régir dans le même temps la politique de l'asile, qui relève du droit humanitaire, et la régulation de l'immigration, qui répond à des considérations tout autres. Insidieusement, l'exécutif laisse germer l'idée que l'attribution du droit d'asile devrait être régulée au même titre que l'immigration, comme si les exilés aujourd'hui bénéficier du statut de réfugié devaient voir leur demande traitée comme celles des requérants venus pour des raisons économiques. Au groupe CRCE, nous nous refusons bien évidemment à procéder à une gradation des misères et des raisons qui poussent les gens à s'arracher à leur terre natale.

afin que les exilés qui formuleront une demande de titre de séjour sur notre territoire puissent bénéficier d'un droit d'asile effectif et indépendant de la politique migratoire, qui relève des compétences de l'administration de la place Beauvau.

de la commission des lois. Puisque beaucoup de nos collègues ont jugé indispensable de s'étendre sur le sujet, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'intervenir à mon tour. Je voudrais vous dire que cette question aurait une véritable importance si les pouvoirs exercés par l'OFPRA étaient discrétionnaires, si l'OFPRA prenait ses décisions sous les ordres d'un ministre. Mais tel n'est pas le cas ! L'Office applique des procédures, que nous sommes d'ailleurs en train de modifier, qui sont de niveau législatif. Il applique également des règles fixées par la Constitution, les conventions internationales et les directives européennes. Vous pourriez décider de rattacher l'OFPRA au ministère de la jeunesse et des sports

vérifier les droits des demandeurs d'asile pour faire en sorte que le taux des décisions annulées par la Cour nationale du droit d'asile

Monsieur le président Bas, permettez-moi de vous dire que je suis complètement en désaccord avec ce que vous venez de dire. Ce sujet n'est pas à prendre à la légère. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse : les salariés de l'OFPRA l'ont eux-mêmes dit lorsqu'ils se sont mis en grève il y a

de rappeler la spécificité des protections internationales que représentent les statuts de réfugié, de protégé subsidiaire et d'apatride, ce que n'assure pas le ministère de l'intérieur.

Heureusement, dans notre pays, l'État est un, et les ministères ne suivent pas des politiques contradictoires.

est passible de sanctions pénales. La convention de Genève et la directive Qualification de 2011 protègent d'ores et déjà les pratiques d'avortement ou de stérilisation forcés, qui peuvent être prises en compte dans la définition de l'appartenance à un certain groupe social.

l'avortement ne peut pas se traiter indépendamment du cadre européen. La définition de la liste des pays sûrs découle en effet directement de la directive Procédures. Or je rappelle que, dans plusieurs États membres de l'Union européenne, qui sont considérés comme des pays sûrs en vertu du protocole « Aznar » annexé au traité d'Amsterdam, l'avortement est interdit ou pénalement réprimé.

Comme l'a rappelé une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013, la seule pénalisation d'une pratique ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution, car il faut que la peine soit effectivement appliquée contre un groupe social et dans des conditions qui s'apparentent à une persécution à l'égard de ce groupe. L'existence d'une infraction pénale n'est pas suffisante pour caractériser une persécution. Pour bénéficier de la protection subsidiaire, il faut ainsi prouver que l'on est exposé dans son pays à un risque de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains et dégradants, ou encore d'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.

qu'une femme meurt d'un avortement clandestin toutes les quatre minutes sur la planète, si ce n'est pas une persécution, je ne sais pas ce que c'est ! Madame la ministre, je ne retirerai pas mon amendement, ce dont vous vous doutiez, j'imagine, et je vous demande d'assumer votre avis défavorable sur cet amendement

et écorne l'image que nous donnons de nous dans le monde. Nous devons rester la flamme de la liberté, des droits des personnes, du respect et de la protection qui leur sont dus.

En attendant, puisqu'il existe une liste de pays sûrs, la France ne doit pas accepter dans cette liste un pays qui condamne des femmes qui ont avorté

paritaire a voté cet amendement « élastique » à l'unanimité. Quand on vit dans un pays où il faut inscrire dans la loi que les femmes militaires auront droit à un uniforme particulier, parce qu'elles sont enceintes,

Le scrutin est ouvert.

Merci